La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener une mission d'information sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de protection de hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquements. Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de sa séance de ce matin.

toutes les personnes qui peuvent apporter un éclairage sur l'affaire communément appelée « affaire Benalla » et, bien au-delà, sur les dysfonctionnements que nous avons constatés sur deux points essentiels : premièrement, la confusion des pouvoirs entre les responsabilités constitutionnelles du Président de la République et celles du Gouvernement dans la mise en oeuvre de la politique de sécurité ; deuxièmement, les difficultés que cette confusion des pouvoirs fait apparaître en ce qui concerne les conditions de mise en oeuvre de la sécurité du Président de la République, qui doit être confiée non pas à des amateurs, mais à des à des professionnels formés, sélectionnés, entraînés et organisés pour assumer cette fonction de protection, dans l'intérêt supérieur de la République. Ces pouvoirs, si vous nous les accordez, nous permettront, d'une part, d'auditionner

qui nous sera indispensable concernant, par exemple, des notes internes de service, utiles pour bien comprendre le fonctionnement de l'État. Je signale que toute personne qui refuserait d'apporter son concours ou qui ferait obstruction à la commission des lois dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation serait passible d'une peine allant jusqu'à deux ans de prison et 7 500 euros

le secrétaire général de la présidence de la République, le préfet de police, un certain nombre de hauts fonctionnaires civils et militaires, les syndicats de la police nationale et toute personne susceptible de nous éclairer. La parole est à M. le président

pas simplement en cause un individu, un lampiste, un « bagagiste », comme l'a dit avec un sens de l'humour consommé M. Castaner ce matin. Elle met en cause nos institutions et, d'abord, l'autorité de l'État. Comment se fait-il qu'un individu déguisé en policier se retrouve au coeur d'une opération de maintien de l'ordre et tabasse des manifestants, au risque d'ailleurs de salir l'honneur de la police nationale Elle blesse aussi le principe d'égalité devant la loi. On a en effet un sentiment de très grande impunité. Alors même que l'Élysée

a été reconnu au moment de la panthéonisation de Simone Veil, tout près d'ici, et au commandement, ou presque, du bus qui ramenait les Bleus jusqu'au Palais de l'Élysée. Il y a donc un problème de fonctionnement de nos institutions. Cette affaire révèle une pratique institutionnelle qui n'est pas acceptable.

debout, sur ses deux pieds, avec un bicamérisme dont on voit bien qu'il assure ici la continuité, notamment, de la République et des pouvoirs, un véritable bicamérisme avec un Sénat en mesure de faire valoir sa responsabilité et ses droits ? La parole est à M. le président

Je ne reviendrai pas, une nouvelle fois, sur la gravité de la crise politique que nous traversons. J'ai eu l'occasion de le faire encore ce matin, par la voie d'un rappel au règlement. Mais il est vrai que des choses se sont passées ce week-end et que l'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était déroulé. De nouveaux éléments sont apparus. Pour moi,

les fait vaciller. J'y vois aussi un lien avec le projet de loi constitutionnelle, dont le débat a été suspendu à l'Assemblée nationale. Si j'ai bien compris,

se conduisent déjà comme des procureurs- ils demandent une commission d'enquête, alors qu'apparemment ils ont déjà toutes les réponses -d'attendre les auditions pour savoir exactement ce qu'il en sera à la fin. Nous verrons bien alors !

La parole est à Mme Maryse

comportement est hautement répréhensible- la justice a été saisie sur ce point -, mais sur des faits de nature politique qui mettent en jeu des questions d'ordre institutionnel. Les faits dont il est question ne peuvent, hélas, que nourrir les populismes et la défiance envers les responsables Je veux également saluer le choix responsable du Sénat de ne s'aligner ni sur le périmètre d'investigation ni sur la méthode retenus par nos collègues députés, mais de s'interroger de façon plus large sur l'exercice de missions de maintien de l'ordre par des personnes extérieures aux forces de sécurité intérieures. S'il le fallait encore, cette décision démontre que notre démocratie a besoin d'un bicamérisme équilibré et fort, assorti de contre-pouvoirs responsables, à même de maintenir le lien de confiance entre nos concitoyens et leurs élus. Dans le contexte de réforme de nos institutions, ce point est d'autant plus fondamental. Cette commission d'enquête permettra au Sénat d'exercer pleinement sa mission de contrôle. Nous souhaitons que ses travaux soient menés dans la plus grande sérénité possible, afin que nos décisions ne soient pas dictées par l'émotion. Pour ces raisons, notre groupe votera évidemment en faveur de la demande de la commission des lois. Très

Territoires. Au nom du président Malhuret, j'exprime le soutien du groupe Les Indépendants à la création de cette commission d'enquête.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Michelle Gréaume, sur l'article. Nous abordons un élément important de ce texte. Très logiquement, et comme cela avait été le cas avec la loi Égalité et citoyenneté, la commission a été au bout d'une certaine logique et d'une volonté farouche depuis maintenant plus de dix ans : enterrer la loi SRU. Cette loi- et il n'est vraiment pas inutile de le rappeler -est un vrai marqueur de notre République sociale et fait consensus depuis Personne jusqu'à présent n'avait osé s'y attaquer tant le symbole est lourd de sens. Aujourd'hui, tout est bon pour y parvenir : il faut laisser plus de temps, alors même que la loi Duflot a déjà accordé cinq années supplémentaires

La majorité sénatoriale nous montre, une fois de plus, sa conception toute particulière du droit au logement et, plus spécialement, du logement social. Le Gouvernement, comme d'autres avant, lui donne de sérieux points d'appui : les dotations aux collectivités sont en berne, les aides à la pierre sont dramatiquement sont dramatiquement basses. Alors que l'État se désengage, le discours de responsabilité adressé aux communes qui doivent respecter les obligations de la loi SRU semble pour certains de plus en plus inacceptable. Nous l'entendons. mes chers collègues, c'est que, sur des constats identiques, nos réponses divergent et nos engagements sont à l'opposé. Nous oeuvrons, pour notre part, en faveur de l'augmentation des aides à la pierre et pour le respect des collectivités par un niveau de dotations qui leur rende une réelle marge de manoeuvre. Nous agissons aussi pour le respect du droit au logement et pour la dignité des personnes. Comment ne pas voir l'urgence de construire davantage de logements sociaux partout, même là où il y en a déjà, quand il en manque près de 2 millions ? Nous ne serons pas complices de ce détricotage de la loi SRU, de cette attaque en règle contre le droit au logement. Nous sommes non pas pour le chacun pour soi, mais pour les solidarités entre les collectivités et entre les citoyens. Construire des logements sociaux, c'est à la fois porter un modèle social de progrès et afficher la volonté politique que soient respectés les droits fondamentaux de chacun, dont celui d'avoir un toit pour se loger.

de participer à l'étalement urbain, mais, par exemple, ... S'il vous plaît ! ...de réhabiliter le parc ancien et d'en changer la destination. Beaucoup de communes s'engagent dans cette direction. C'est donc bien un objectif utile, plus nécessaire que jamais, alors que la crise du logement se manifeste de manière accrue.

Les intercommunalités sont les chefs de file reconnus des politiques locales de l'habitat menées sur les territoires, au travers de la mise en oeuvre de PLH [ ...], dans le respect de l'exigence de mixité et de répartition équilibrée du parc social

Il semble que la mise à mal de quelques avancées sociales soit un objectif de ce gouvernement et de la majorité sénatoriale. Si ces avancées sociales ne possédaient plus aucune vertu, nous pourrions le comprendre ... Pour quelle raison la loi SRU est-elle considérée comme une telle avancée ? Peut-être parce que, malgré les critiques qui lui sont souvent adressées sur son manque d'efficacité, elle a tout de même permis de construire plus de 600 000 logements en Peut-être aussi parce qu'elle poursuit l'objectif de créer un équilibre social entre les territoires. Enfin, parce que cette loi, comme l'avait rappelé l'abbé Pierre à l'Assemblée nationale le 26 janvier 2006 lorsqu'elle avait été mise en danger- déjà -par la droite, relève de l'honneur de la France, en ce sens qu'elle offre une certaine protection aux plus précaires. Cet article est la contrepartie de l'article 29, qui vise à céder le parc locatif social français à des personnes privées. L'objectif n'est autre que la vente de logements sociaux. La loi SRU est en travers de votre chemin, alors vous voulez l'abattre ! L'article 46 étend de cinq à dix ans la durée pendant laquelle les logements sociaux vendus resteront comptabilisés dans les « quotas SRU », et ce dans l'objectif annoncé de lever les réticences à la vente de ces logements sociaux en accordant aux communes un délai pour reconstituer leur stock. Or cet allongement du délai permettra en fait aux communes, particulièrement à certaines communes carencées, qui ne respectent pas leurs obligations, de tricher et d'éviter un effort de construction. Alors que 2 millions de personnes en France attentent un logement, la vente dans ces communes carencées est une aberration. La commission a largement aggravé cette disposition en détricotant méthodiquement l'article 55 de la loi SRU. Qu'y a-t-il derrière ces dispositions ? Plus de profits pour le privé, et un moyen d'éviter la mixité et de favoriser l'entre soi dans certaines communes ou certains quartiers. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même : ce sont toujours les plus précaires qui en subiront les dommages. Comment en est-on arrivé à privilégier ceux qui ont le moins besoin de privilèges ? », demandait l'abbé Pierre en février 2006. Avec ce projet de loi, comme avec presque tous ceux que nous avons examinés ici depuis quelques mois, quelques pas supplémentaires ont été franchis dans cette direction. Je vous remercie

l'article. Dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, la démolition de logements sociaux peut conduire à une chute importante du nombre de ces logements dans la commune qui bénéficie du programme de l'ANRU. Le temps de reconstituer l'offre, la commune peut se retrouver dans une situation de déficit de logements par rapport aux objectifs de la loi SRU. SRU. Elle pourrait alors être soumise à un prélèvement annuel sur ses ressources fiscales, ou voir celui-ci fortement augmenter, alors même qu'elle est mobilisée pour le financement d'importants investissements dans le cadre du programme ANRU. Afin de laisser le temps à la commune de reconstituer une offre de logements sociaux, je propose que les logements démolis continuent à être comptabilisés, au titre de l'article 55 de la loi SRU, pendant une période de dix ans à compter de leur démolition, à condition que la reconstitution de l'offre de logements sociaux en compensation des logements démolis soit identifiée. Pour avoir été maire d'une commune où ont été démolis de nombreux logements sociaux,

Pour des raisons souvent historiques, ces communes- pas qu'en Seine-Saint-Denis, je le redis -n'ont pas forcément un taux de logement social élevé. Pour autant, elles accueillent des ménages pauvres en nombre.

Qu'il s'agisse des amendements sur l'article 46 ou des articles additionnels après l'article 46, je suis effaré, mais pas surpris, de voir la majorité sénatoriale faire totalement fi des 4 millions de personnes mal logées dans ce pays. En comptabilisant dans les 25 % de logements sociaux des logements provisoires, tels que les centres d'hébergement, les logements d'urgence, les PSLA, en permettant aux communes ayant 15 % de logements sociaux de renégocier le calendrier pour atteindre 25 % sans cadrage dans le temps, en mutualisant à l'échelon des EPCI le reste à construire des logements sociaux par les communes, vous vous attaquez sans ambages à la mixité sociale, vous faites de la dérogation la règle, vous dévitalisez avec méthode la loi SRU, en opposition à toute logique de justice et de bon sens économique. Avec ces dérogations, vous allez engendrer une concentration de la construction dans certaines villes en dédouanant les autres de leur devoir de mixité sociale. La loi SRU est un puissant outil de construction de logements sociaux sur les territoires, on l'a déjà dit, et de mixité sociale. Avec mon groupe, nous défendrons une loi pragmatique, qui permet de construire la moitié des logements sociaux neufs du pays dans les communes qui en manquent cruellement et qui, bien souvent, y sont réticentes. Rappelons à quoi sert cette loi : à organiser une politique de production harmonieuse de logements sociaux pour les plus modestes, qui n'ont pas la possibilité de se loger. Comment pouvons-nous revenir sur cette loi qui est en quelque sorte un acquis social ?

Permettez-moi de prendre, pour conclure, l'exemple de mon département, les Hauts-de-Seine. Si, comme vous le souhaitez avec l'amendement de Mme la rapporteur, nous faisons sortir les communes de moins de 3 500 habitants en Île-de-France du dispositif SRU, une ville qui ne connaît pas les plus grandes difficultés financières, Marnes-la-Coquette, n'aura plus à répondre à son engagement de construction de logements sociaux, alors même que nous sommes dans une zone tendue pour les logements. Comment peut-on se permettre, quand 70 % des Franciliens sont éligibles au logement social, d'avoir, d'un côté, des poches de privilégiés et, de l'autre, des poches de défavorisés ? La mixité sociale est le ciment de notre République, et chacun doit en prendre sa part dans la lutte contre la ségrégation sociale. La parole est à Mme Viviane Artigalas,

ont pour objectif la disparition de l'article 55 de la loi SRU et, donc, des quelque 700 000 logements sociaux attendus d'ici à 2025 dans les communes carencées et déficitaires. Le calendrier, le taux, la mutualisation, le financement, le nombre de logements décomptés : tout est encore remis en cause ! Pourtant, la loi SRU est une loi « socle » de notre République, un texte fondateur en matière de mixité sociale. Nous avons déjà eu un débat important il y a moins de deux ans au travers de la loi Égalité et citoyenneté. Cette loi majeure du précédent quinquennat a consolidé le périmètre d'application du dispositif SRU pour le rendre plus cohérent avec la réalité du terrain. Un certain nombre de communes peuvent en effet sortir du dispositif, notamment lorsque la demande de logements n'est pas suffisante ou lorsque les communes sont insuffisamment desservies par les transports. La loi a également renforcé les moyens opposables aux communes qui s'exonèrent de l'effort national de solidarité. C'est essentiel Il faut continuer la pression sur les territoires dits tendus, où la demande de logement est très importante. La loi SRU répond à des logiques de solidarité qui doivent s'imposer à toutes et tous. Nous nous opposerons

Le présent projet de loi n'a pas pour dessein la remise en cause de la loi SRU. Il me semble d'ailleurs que le Gouvernement a démontré, depuis maintenant plus d'un an, son ferme attachement à une loi qu'il juge bonne, en ce qu'elle favorise la mixité sociale. part cependant d'un constat : les communes hésitent fortement à donner un avis favorable à la vente de logements sociaux à leurs occupants- ayant été maire d'une commune de 20 000 habitants, je peux attester de cette difficulté -, de crainte de ne pas parvenir à reconstituer à temps le parc de logements sociaux correspondants, et donc d'être pénalisées. Pourtant, faciliter la vente de ces logements à leurs occupants est un moyen de rendre accessible la propriété pour les ménages les plus modestes, de renforcer la mixité sociale que nous appelons tous de nos voeux et de dégager des ressources pour les organismes d'HLM afin qu'ils puissent rénover leur parc de logements et en construire de nouveaux. Allonger de cinq à dix ans la durée pendant laquelle des logements sociaux vendus à leurs occupants seront pris en compte dans le quota fixé par la loi SRU est un moyen d'apporter une réponse pragmatique et efficace à cet enjeu majeur, qui concerne en premier lieu les ménages les plus modestes. Enfin, j'aimerais mettre un terme aux inquiétudes que l'on a pu entendre jusqu'ici, légitimes pour certaines d'entre elles, sans doute moins, et il faut le regretter, pour d'autres. Mes chers collègues, il va de soi que l'allongement proposé est strictement encadré : il ne pourra bénéficier qu'aux ventes réalisées au bénéfice du locataire occupant, et en aucun cas aux ventes en bloc.

Ainsi, sur la période 2011-2013, elle a réalisé ses objectifs à hauteur de 208 % et, sur la période 2014-2016, alors même que les dernières données ne sont pas consolidées, à hauteur de 161

à plusieurs dizaines, voire à des centaines de kilomètres et de prendre le train tous les jours pour venir travailler à Paris ? En matière de politique du logement, il est plus que nécessaire de créer une continuité entre le logement social, le logement intermédiaire et le logement dans le parc privé.

des accords possibles ou des fongibilités ? Il faut en effet une disponibilité foncière en même temps qu'un certain nombre d'équipements susceptibles de répondre aux besoins de mobilité et de proximité des équipements publics

que les territoires qui ont des responsabilités éminentes dans ce domaine puissent conduire graduellement et avec efficacité les programmes qu'ils veulent développer ensemble.

Il n'est nullement dans les intentions du Gouvernement de mettre à mal et d'abattre cette loi, dont je dis depuis le début des débats à l'Assemblée nationale et même avant, puisque j'ai eu à répondre

Il y a un corpus qu'il convient de conserver, parce qu'il a fait ses preuves. Cette loi a montré son utilité en termes d'accélération de la construction de logements sociaux. Cela étant, au fil des ans,

qu'elles ne respectaient pas leurs obligations légales et devaient produire des logements sociaux pour rattraper leur retard. 711 communes ont respecté le taux légal de logement social applicable, 649 communes n'ont pas atteint les objectifs de rattrapage triennaux fixés sur la

le renforcement des sanctions initialement envisagées par les préfets dans les communes les plus récalcitrantes. Je n'ai pas hésité à le faire. Si le Gouvernement avait eu l'intention de mettre à bas la loi SRU, je n'aurais pas écrit

Madame la rapporteur, vous avez parlé

enterrer, inhumer ou faire disparaître la loi SRU. L'article 55 de la loi SRU a été un déclencheur, comme l'a dit Valérie Létard, qui a permis de faire prendre conscience à un certain nombre de territoires de la nécessité de construire

les logements objets d'un bail réel solidaire, parce que l'occupant de ce logement est soumis à des conditions de ressources ; troisièmement, sur proposition de la commission des lois, comme l'a rappelé Marc-Philippe Daubresse, les places d'hébergement d'urgence, conformément à ce qui a été voté dans

et 2031. Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, la réforme territoriale est passée par là, en favorisant le regroupement des communes ou le développement des EPCI, qui a conduit bon nombre de communes à être désormais soumises aux dispositions de la loi SRU. Je pense plus particulièrement aux communes nouvelles et aux communes entrantes, qui n'ont été intégrées au dispositif qu'à partir du 1 janvier

déterminerait le nombre de triennats nécessaires pour atteindre ce taux de 25 %, ainsi que les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux que la commune s'engage à respecter

dans lesquelles le taux de pauvreté des ménages dépasse 25 % dans le parc locatif. Cette proposition, si elle amorce un changement de paradigme, nous semble suffisamment encadrée

pour permettre aux maires de réaliser leurs obligations en matière de construction de logements sociaux à hauteur de 25 %, mais dans de bien meilleures conditions qu'actuellement. Il ne s'agit en aucun cas, je le répète, et nous nous sommes tous engagés sur ce point, d'exonérer les maires de leurs obligations. Les maires sont responsables, et ils continueront à s'inscrire dans la volonté de construire du logement social. C'est la raison pour laquelle,

de même, car confrontées à des réalités qui rendent totalement impossible le fait de construire des logements sociaux dans les proportions que nous décidons. Sinon, nous aurons un faux débat. Il ne s'agit pas de faire l'historique des votes des uns et des autres.

de manière considérable, alors que celle-ci a déjà fait ses preuves. Pourquoi revenir sur un dispositif législatif, qui, malgré ses quelques imperfections, favorise la construction de logements sociaux ?

Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les raisons que j'ai précédemment expliquées. Je rebondirai très rapidement sur la question des exemptions,

même pour les communes qui ont toujours, jusque-là, respecté leurs engagements triennaux. Je ne vous parle pas des maires qui ne veulent rien faire, ni de ceux dont les communes ont déjà été carencées. Je vous parle des maires dont les communes, depuis 2000, n'ont jamais été carencées, ont toujours tenu les objectifs triennaux et qui vont droit dans le mur.

Le maire et les élus sont responsables devant leurs électeurs. Le maire, les élus et leurs équipes sont responsables pour aménager les communes et pour loger leurs habitants. Du Du fait du vieillissement de la population, de la décohabitation, des divorces, il faut construire partout, notamment en zone tendue, pour tout simplement maintenir la population. Dans leur immense

et rendue pragmatique, afin de continuer à accompagner les maires dans leur obligation de construire 25 % de logements sociaux, mais d'une façon réaliste. Sur l'amendement du Gouvernement, l'avis est également défavorable, bien entendu.

Par cet amendement, nous proposons d'appliquer le calcul du taux de logements sociaux à l'échelle de l'agglomération ou de l'EPCI, et non de chaque commune.

La loi SRU a permis de répondre efficacement aux impératifs de création de logements depuis sa promulgation en 2000. Par l'intermédiaire du plan local d'urbanisme, de nombreuses communes se sont fixé des objectifs plus ambitieux de création de logements à vocation sociale. Les dispositions de cette loi doivent donc être maintenues pour continuer de répondre aux enjeux de logement et d'aménagement du territoire dans notre pays. Toutefois, il apparaît, dans un certain nombre de cas, que l'application de la loi SRU n'est pas optimale et entraîne des incohérences quant à l'articulation entre les différents documents d'urbanisme que doivent respecter les communes. Ainsi, plusieurs communes en France se trouvent être rattachées, pour l'application de la loi SRU, à des agglomérations autres que celles dont elles dépendent pour l'établissement du schéma de cohérence territoriale. Pour une plus grande cohérence Pour une plus grande cohérence dans l'application de la loi et la réalisation des plans locaux d'urbanisme, des plans locaux de l'habitat et des schémas de cohérence territoriale, nous proposons de préciser qu'une commune ne peut être rattachée, pour l'application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de qu'à une agglomération dont la majorité des communes se trouvent dans le périmètre du même schéma de cohérence territoriale que la commune concernée. Cela paraît l'évidence

dans le calcul du taux SRU, les logements intermédiaires. Ces amendements visent à les retirer du nombre de logements total du parc, de manière à ne pas désinciter les maires à construire et à aider au financement de ce type de logements, qui répond aux besoins d'une partie de la population, celle qui est trop riche pour être dans le parc HLM et, en même temps, trop pauvre pour se loger dans le parc privé. Je profite du temps qui m'est imparti pour

du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, qui tient compte de la servitude d'utilité publique liée à la présence du domaine national du château de Versailles sur notre commune,

et aux logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Elle a également pris en compte les places d'hébergement en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, en centres d'hébergement

visant à intégrer dans le décompte des quotas de logements sociaux imposés aux communes au titre de la loi SRU les structures d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile et les centres d'hébergement provisoire destinés aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection L'hébergement des demandeurs d'asile est une obligation morale, mais il ne faut pas tout mélanger. Les politiques d'asile et de protection des demandeurs ne sont pas des politiques d'accès au logement. L'objectif de la loi SRU est de maintenir au sein de l'offre de logements

d'un PSLA ou les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Une telle disposition altère à nos yeux l'objectif même de la loi SRU, à savoir la présence dans l'ensemble des communes d'un taux de logement social suffisant pour répondre à la demande.

part, nous ne sommes pas favorables à cette intégration. Nous préférons en rester à l'objectif de la loi SRU, d'autant que le dispositif prévu

n'entraîne pas la perte des logements construits dans le cadre des contrats intercommunaux de mixité sociale, qui restent réputés construits sur le territoire. Ce dispositif a fait l'objet

285 rectifié tend à intégrer à l'inventaire des logements sociaux SRU les places créées dans des maisons d'enfants à caractère social. Nous y sommes défavorables.

et à la citoyenneté a recadré les possibilités de recours à cette mutualisation : le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif triennal. Quelles sont les raisons de ce recadrage ? Le dispositif a été trop souvent détourné : les communes l'utilisaient pour diminuer leur objectif de production et éviter la carence, sans pour autant mettre en oeuvre une démarche volontariste en vue de rattraper le retard. Il faut également rappeler que seule une trentaine d'EPCI sur 211 dotés de la compétence logement et d'un PLH exécutoire utilisaient ce dispositif de mutualisation. Par la décision rendue par la juridiction administrative de Cergy-Pontoise concernant la ville d'Asnières-sur-Seine, dont j'ai parlé la semaine dernière, les juges ont rejeté la demande du préfet, considérant que le programme attaqué, qui ne comportait pas de logements sociaux, se situait à proximité immédiate du secteur des Hauts d'Asnières, un quartier de la ville dont le pourcentage de logements sociaux reste voisin de 70 %.

de manière à ne pas dispenser complètement les communes dont 35 % ou 40 % du territoire est pénalisé par des inconstructibilités, mais à ne pas non plus leur imposer la totalité de l'obligation, ce qui, avec une telle neutralisation de territoire urbanisable, se révèle

Fouché. Nous proposons d'inclure les résidences-services destinées aux personnes âgées ou aux personnes handicapées parmi les logements locatifs sociaux pris en compte pour l'application de l'article 55 de la loi SRU dans les mêmes conditions que les logements-foyers de personnes âgées et de personnes handicapées, afin de favoriser leur développement et de reconnaître leur apport à la mixité sociale. les résidences-services, définies à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation, permettent, dans de nombreux territoires, de favoriser la mixité sociale.

En outre, les résidences-services constituent souvent une solution de maintien à domicile adaptée aux besoins de nombreuses personnes âgées ou handicapées, en cohérence avec l'ambition qui sous-tendait la loi d'adaptation

voyage. Ces aires entrent dans le champ des hébergements sociaux, puisque ce sont des lieux de séjour pour des personnes en situation de précarité qui peuvent y rester plusieurs mois, voire plusieurs années. De plus, ces aires représentent un coût non négligeable pour les collectivités locales qui en ont la charge. Enfin, l'intégration des aires d'accueil dans les quotas de logements sociaux serait logique, puisque les dépenses, notamment foncières, engagées par une commune pour la création de ces aires peuvent déjà être déduites des pénalités SRU.

de Cidrac. Cet amendement vise à introduire dans la comptabilité des logements sociaux les résidences hôtelières à vocation sociale et les logements dans les hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté.

Les missions des CCAS sont variées et incluent souvent des actions d'insertion pour les personnes connaissant des difficultés financières. À cette fin, les CCAS mettent des logements en location. Le présent amendement vise à inclure ces logements dans le quota de 25 % de logements sociaux prévu par la loi SRU.

il est proposé que les logements sociaux vendus continuent d'être comptabilisés comme tels jusqu'à dix ans après la vente. Cela vient comme le corollaire de la volonté affichée par le Gouvernement d'encourager la vente des HLM. Rusé, le Gouvernement invente la « SRU fantôme », en permettant, par un simple jeu d'écriture, de diminuer le nombre de logements sociaux dans une commune sans que cela se reflète dans le pourcentage imposé par la loi SRU. On aboutirait ainsi à une sorte de persistance rétinienne du respect de la loi SRU, celui qui, ayant regardé trop longtemps le soleil en face, continue de le voir devant ses yeux plusieurs minutes après les avoir fermés. De plus, cette mesure profitera en premier lieu aux communes où les prix de l'immobilier sont le plus élevés, car c'est dans ces villes que les ventes de logements sociaux ont le plus de chance d'aboutir. Les loyers étant corrélés au prix de vente des logements, on comprend bien que des personnes ou des entreprises souhaitant investir dans l'achat de logements sociaux le feront dans des villes permettant de bons retours sur investissement. Ces villes-

Le projet de loi étend de cinq à dix ans la durée de comptabilisation au titre de la loi SRU des logements sociaux vendus à leurs locataires. Cette mesure a vocation à encourager les communes à vendre leur patrimoine, en leur évitant de perdre le bénéfice des efforts réalisés pour augmenter le parc de logements sociaux sur leur territoire. Dans les zones tendues, compte tenu de la rareté des possibilités foncières, la vente de logements sociaux sera difficilement compensée par la création d'autres logements sociaux. En même temps, faut-il rappeler que les zones tendues manquent cruellement de logements abordables adaptés aux ressources et aux besoins des Français ?

situés dans les zones où a été instituée la taxe sur les logements vacants. Il convient en effet d'amener les bailleurs sociaux soit à limiter la vente de leurs logements, soit à renouveler leur offre locative, afin de ne pas diminuer le volume de logements sociaux effectivement disponibles et de ne pas pénaliser ainsi encore plus les demandeurs de logement social, particulièrement nombreux dans ces zones en forte tension. Quel

Schmitz, pour présenter l'amendement n° 246. Si les communes ont à respecter la règle des 25 % de logements sociaux à l'horizon 2025 en application de la loi SRU, l'État devrait également s'appliquer cette règle en tant que propriétaire d'un parc immobilier. C'est une question récurrente que M. le ministre connaît bien. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, et l'on aboutit même à une véritable double peine- le mot n'est pas trop fort -dans les communes où l'État possède un parc immobilier non conventionné très important. Vous ne serez pas surpris d'apprendre, monsieur le ministre, que tel est le cas de la ville de Versailles. Non seulement ces logements ne sont pas considérés comme des logements sociaux, mais leur prise en compte dégrade de surcroît le ratio de la commune. Rappelons le mode de calcul que tout un chacun connaît au sein de la Haute Assemblée : au numérateur figurent les logements conventionnés, au dénominateur, la totalité des résidences principales de la commune. En conséquence, les communes disposant d'un parc important de logements de fonction propriété de l'État ou de ses établissements publics -en l'espèce, le château de Versailles -sont fortement pénalisées. ces logements-notamment les casernes militaires ou de gendarmerie -ne sont pas comptabilisés au numérateur, car non conventionnés, mais de surcroît ils augmentent le dénominateur, car ils sont considérés comme des résidences principales.

deux fois sanctionnées financièrement du fait même que l'État ne s'applique pas à lui-même, en tant que propriétaire, la disposition légale de quota minimal de logements sociaux. Cet amendement, que je trouve frappé du sceau du bon sens, vise donc à soustraire les logements de fonction propriétés de l'État et de ses établissements publics du décompte du total des résidences principales, sans pour autant les compter comme des logements sociaux. La parole

Valérie Létard, pour explication de vote.

pour les gouvernements qui lui succéderont, l'évolution du département de la Seine-Saint-Denis est devenue un problème d'État. Absolument

lors, plusieurs dispositions législatives sont venues simplifier, consolider ou stimuler les projets de regroupement. Toutefois, la fusion des communes rurales est parfois freinée

sociaux, ou 20 % si le taux de logements sociaux est inférieur à 10 %. En outre, la part des logements financés par les prêts locatifs aidés d'intégration, les PLAI, doit être au moins égale à 30 %. Nous proposons d'aller plus loin en renforçant la proportion de logements financés en PLAI, qui sont les plus accessibles aux ménages en difficulté, pour la porter à 50 % et en réduisant à 10 % la proportion de logements financés en PLS, dont les niveaux de loyer sont en décalage par rapport aux capacités contributives de la majorité des demandeurs. Pour bien comprendre cette différenciation, il faut savoir que, aujourd'hui, plus de 70 % du patrimoine social est financé des PLS. Ils sont donc très largement majoritaires dans l'offre de logement social, alors même que leurs loyers ne sont pas en adéquation avec les ressources En effet, selon une étude réalisée par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, en 2012, 66 % des nouveaux entrants dans le parc social remplissent les conditions de ressources pour accéder aux logements PLAI et 39 % de l'offre locative sociale présente des niveaux de loyers incompatibles avec les plafonds pris en compte dans le calcul des aides au logement.

de la construction de logements locatifs sociaux destinés à assurer la diversité de l'habitat et à renforcer la mixité sociale. Cela fait donc plus de dix-sept ans, mes chers collègues, que des élus et décideurs de toutes appartenances politiques, même parfois opposés par principe à la prétendue « prolifération » des logements sociaux, mettent en oeuvre les dispositifs de la loi SRU, répondant par là même autant aux exigences du texte qu'aux besoins des populations. Comme chacun le sait, l'action en matière d'habitat et de logement se déroule de plus en plus dans le cadre intercommunal et la diversité des réponses apportées à la problématique du logement recouvre bien souvent des expérimentations positives ou des choix innovants et originaux. Devrions-nous donc, comme nous y invite cet article, interrompre les processus engagés qui visent parfois à réaliser quelques opérations, souvent à « taille humaine », de logement locatif social dans des communes où l'on ne connaissait jusque-là que l'habitat rural ancien et le lotissement pavillonnaire, corollaire de l'étalement urbain Extraire les communes d'Île-de-France de 1 500 à 3 500 habitants du champ d'application de la loi SRU, c'est d'abord rompre les logiques intercommunales à l'oeuvre : regardez l'état de la carte intercommunale francilienne. Ainsi, la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, composée de soixante-treize communes des Yvelines, qui exerce, de fait, la compétence « programme local de l'habitat-politique du logement-lutte contre l'habitat insalubre

Les structures intercommunales franciliennes participent bien souvent, notamment dans les départements de la grande couronne, à cette mixité entre véritables villes et villages en partie urbanisés. Depuis longtemps déjà, le logement social n'y est plus synonyme

présenter l'amendement n° 585. La commission des affaires économiques a estimé que la différence de traitement entre les communes franciliennes, soumises à l'article 55 de la loi SRU à partir de 1 500 habitants, et les autres communes de France, assujetties à ce dispositif à partir de 3 500 habitants, ne se justifiait plus.

et à la citoyenneté a apporté de la souplesse grâce à un recentrage du dispositif SRU sur les territoires où la demande de logement social est avérée, tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou, en tout cas, bien desservis par les transports en commun. En contrepartie de ces ajustements, une contribution rigoureuse à l'effort de construction de logements sociaux est attendue. La commission des affaires économiques a adopté des évolutions qui conduisent à reporter la réalisation des objectifs de 20 % ou de 25 a également prévu un calendrier spécifique de rattrapage s'étalant sur une trentaine d'années pour les communes nouvellement soumises à la loi SRU, à la suite des regroupements opérés dans le cadre de la réforme territoriale. Une grande majorité des villes ont déjà dépassé les objectifs fixés pour 2025, d'autres sont en train de les atteindre. La question est de savoir pourquoi certaines communes ont décidé, depuis 2001, de ne pas appliquer la loi.

Le quatrième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que le prélèvement effectué sur les communes qui ne respectent pas les objectifs de proportion de logements sociaux de l'article 55 de la loi SRU est diminué des dépenses exposées pour l'atteindre. Le présent amendement vise à ce que ce prélèvement soit également diminué des dépenses qui auraient été exposées en l'absence du retard causé par les recours déposés contre le ou les permis de construire. En effet, il apparaît que, dans le cas où les recours causent des retards, les communes de bonne foi peuvent se retrouver prélevées pour des raisons indépendantes de leur volonté, alors qu'elles sont engagées dans un processus de mise en conformité avec les objectifs de la loi SRU. Le présent amendement vise à éviter la fraude à la loi concernant cette nouvelle disposition, en prévoyant que celle-ci ne peut être utilisée afin de se soustraire au prélèvement ou pour créer des conditions permettant de se soustraire au prélèvement.

qui déterminerait le nombre de triennats nécessaires pour atteindre le taux de 25 % de logements sociaux, à une échéance à définir avec le préfet. La commission réduit de ce fait le dispositif de la loi SRU à une simple contractualisation locale d'objectifs et de moyens, sans cadrage national cohérent, transparent et homogène. Cette expérimentation n'est pas à même de garantir les objectifs de mixité sociale dans toutes les communes du territoire où la tension du marché locatif est très forte. On ne combattra pas les ghettos si on ne construit pas rapidement du logement social bien réparti.